La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la consultation du Parlement sur la nomination de membres français dans certaines institutions européennes, présentée par M. Jean François Rapin

remerciements à nos rapporteurs, Agnès Canayer pour la commission des lois et Pascal Allizard, qui est représenté ce soir par

certains au travers de leur commission des affaires européennes, d’autres au travers de commissions spéciales. Neuf parlements participent au processus de désignation du candidat à la Cour des comptes européenne et onze au processus de nomination des candidats au Tribunal et à la Cour de justice de que le groupe de travail sénatorial sur la réforme des institutions présidé par Gérard Larcher avait également, parmi les propositions formulées dans son rapport de mai 2024 pour redynamiser la démocratie, appelé à davantage associer le Parlement à

article 1, une audition obligatoire par la commission des affaires européennes de chaque assemblée du Parlement, ouverte à l’ensemble des membres des commissions permanentes, du candidat national pressenti au poste de commissaire européen.

L’article 2, dans son état initial, précisait les modalités d’organisation d’une audition obligatoire du candidat national pressenti au poste de membre de la Cour des comptes européenne. Le dispositif prévoit que le candidat sera entendu

l’audition obligatoire des candidats aux fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne et de juge du Tribunal de l’Union européenne. Je l’amenderai de la même façon pour clarifier la procédure Je veux souligner qu’une telle démarche n’interfère en rien avec les négociations sur les portefeuilles des commissaires européens et que le dispositif proposé n’est en rien contraire aux dispositions des traités européens. pour l’état des lieux. Sur un plan plus politique, j’entends déjà les récriminations, celles du Gouvernement, en particulier, quant au fait que ces nominations relèvent du domaine réservé. Peut on considérer aujourd’hui, monsieur le ministre, que les affaires européennes n’ont pas évolué depuis l’écriture des textes européens et de notre Constitution ? N’y a t il pas, à ce jour, une intrication forte entre le domaine réservé du Président de la République, les orientations du Gouvernement et la parole du Parlement national sur les institutions européennes ? Vous qui étiez Vous qui étiez déjà ministre chargé des affaires européennes sous le gouvernement Barnier, vous étiez, et j’avais trouvé cela significatif, le seul ministre à avoir deux fois votre photo sur l’organigramme du Gouvernement rattachement au Quai d’Orsay et une fois sous l’autorité directe du Premier ministre. N’était ce pas significatif de ce pouvoir partagé ? Et, malgré la séparation des pouvoirs, pourquoi le Parlement n’aurait il pas son mot à dire aussi, par ailleurs, les procès en inconstitutionnalité. Croyez vous que le président de la commission des affaires européennes, seule commission constitutionnelle, voudrait trahir ou détourner la Constitution ?

On a inventé, en sus de la démocratie représentative, la démocratie participative. Quant à moi, je suis pour la démocratie tout court. Ce texte, monsieur le ministre, en est un exemple. La parole

vise à assurer un rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif et le Parlement pour ce qui est de la nomination à certaines fonctions européennes ; c’est à une anomalie démocratique de ce qui se passe dans d’autres États membres de l’Union européenne, la désignation des candidats à certaines fonctions éminentes au sein des institutions européennes échappe totalement au regard du Parlement. Si la Si la séparation des pouvoirs est un principe cardinal de nos institutions, elle ne saurait exclure une collaboration entre le Parlement et l’exécutif, dès lors que l’objectif est celui d’une plus grande transparence démocratique. Au regard de la place croissante qu’occupe le droit de l’Union européenne dans notre ordre juridique, au regard aussi des conséquences qu’emportent certaines décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la Commission européenne, l’absence d’association du Parlement à la désignation des candidats est regrettable. Le feuilleton de la désignation du nouveau commissaire européen, l’été dernier, a démontré les limites du silence de notre droit positif, qui laisse aux « autorités nationales » toute liberté pour choisir le candidat français. La désignation de Thierry Breton au mois de juillet, puis son remplacement dans la précipitation par Stéphane Séjourné en septembre, sans aucune concertation et par simple communiqué de presse, ont pu légitimement susciter certaines interrogations. Cette proposition de loi agit comme un révélateur de l’opacité des conditions de cette désignation et de l’absence du Parlement français dans le processus. Cette anomalie avait d’ailleurs déjà été révélée par les travaux du Sénat. La proposition de loi prévoit donc de soumettre à une audition préalable les candidats pressentis pour occuper les fonctions de commissaire européen – c’est l’article 1 –, de membre de la Cour des comptes européenne – c’est l’article 2 – et de juge ou d’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne En effet, si les fonctions visées sont exercées au sein des institutions de l’Union européenne, le choix des candidats est une question purement nationale. Les traités européens laissent en effet libre choix aux États membres de déterminer comment les candidats sont proposés et surtout par qui. l’autorité compétente, l’usage récent semble réserver au Président de la République le soin d’annoncer par courrier le choix des autorités françaises, et le rôle du Premier ministre n’est absolument pas clair.

En effet, la participation de la France à l’Union européenne et l’exercice en commun des politiques publiques relèvent avant tout de la conduite de la politique de la Nation, que l’article 20 de la Constitution confie au Premier ministre, responsable devant le Parlement.

le pouvoir de nomination du Président de la République ou du Premier ministre à une simple audition par le Parlement, sauf si une disposition constitutionnelle le prévoit. En l’espèce, la désignation des candidats, qui participe de la politique européenne de la France, est non pas une nomination à proprement parler, mais une simple proposition de nomination. En effet, les nominations sont prononcées par les instances européennes, non par les autorités françaises, qui n’ont qu’un simple pouvoir de proposition. En outre, l’avis qui serait rendu

ou encore de fragiliser la posture de la France dans les négociations sur l’étendue de son portefeuille. L’actualité montre d’ailleurs que le fait du prince ne garantit pas l’influence de notre pays, particulièrement si le candidat est perçu comme étant celui du Président de la République et non celui de la France. Au contraire, l’avis favorable des commissions compétentes ne pourrait que renforcer la position de la France et celle du candidat. En outre, la consultation du Parlement conduirait également l’exécutif à être particulièrement vigilant sur la qualité et l’expérience des candidats qu’il envisagerait de désigner.

en témoignent les décisions de la CJUE relatives au temps de travail des militaires ou à la conservation des données personnelles. Le Parlement a donc toute sa place. Ces auditions permettraient notamment de connaître la vision des candidats et de vérifier leur aptitude à réfléchir à l’articulation des systèmes juridiques européens européens et nationaux. L’association du Parlement à ces désignations est non seulement légitime, mais elle constitue une véritable nécessité démocratique. Mes chers collègues, il ne nous est pas donné tous les jours de défendre les droits et le rôle du Parlement. Ce texte nous en offre l’occasion et il nous appartient de la saisir. C’est pourquoi la commission des lois a émis un avis favorable sur l’adoption de cette proposition de loi, modifiée par les amendements présentés par Jean

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai ce soir la voix du rapporteur pour avis Pascal Allizard, pour qui la proposition de loi du président Jean François Rapin soulève des questions d’un vif intérêt juridique et d’une grande importance politique. Ses trois articles prévoient de faire précéder d’une audition parlementaire le choix des candidats français destinés à siéger à la Commission européenne, à la Cour des comptes européenne et dans les institutions judiciaires européennes. Mieux partager le pouvoir de nomination pour rééquilibrer les institutions a été un objectif partagé dès avant la réforme de 2008.

Dans ce contexte, nul ne comprendrait qu’une fonction aussi importante que celle de commissaire européen reste l’objet de tractations de couloir au sommet de l’État. Le secrétariat général du Gouvernement (SGG) estime toutefois que la jurisprudence du Conseil constitutionnel fait obstacle à cette initiative. Le principe de la séparation des pouvoirs empêche effet, selon le juge, que le pouvoir de nomination par une autorité administrative soit subordonné à une audition parlementaire. L’application de cette jurisprudence au choix du commissaire européen n’est cependant pas évidente. D’abord, quelle est, au juste, la procédure en cause ? Nos textes n’en disent rien et la doctrine à peine davantage.

dernier, la désignation des candidats aux institutions européennes est « assimilable à une nomination », dont la compétence de principe est conférée par la Constitution à l’exécutif seul. Notre commission des affaires étrangères n’est certes pas compétente au fond en matière constitutionnelle, mais elle l’est sur les questions européennes. Cela tombe bien, car c’est dans le traité sur l’Union européenne que se trouve la base juridique pertinente. Son article 17 prévoit que le Conseil propose un collège de commissaires à l’approbation du Parlement européen sur la base des « suggestions faites par les États membres », avant nomination par le Conseil européen. Si « suggestion » valait nomination, la candidature de Mme Sylvie Goulard, par exemple, n’aurait pas été rejetée par le Parlement européen en 2019. Le terme de « suggestion » est même si peu précis que la présidente réélue von der Leyen s’est crue autorisée, cet été, à exiger de l’Irlande et de la Bulgarie qu’elles proposent chacune une liste d’au moins deux candidats, dont un homme et une femme. La décision des États emporte donc trop peu d’effets prévisibles pour qu’on puisse la qualifier d’acte de nomination au sens du droit administratif français. Mais l’emploi que le candidat est appelé à occuper n’entre pas non plus facilement dans nos cases juridiques habituelles. Le Président de la République a un pouvoir général de nomination « aux emplois civils et militaires de l’État et le Premier ministre un pouvoir subsidiaire de nomination « aux emplois civils et militaires », car c’est lui qui « dirige l’action du Gouvernement », lequel « détermine et conduit la politique de la Nation Le traité précise cependant que la Commission européenne « promeut l’intérêt général de l’Union », qu’elle exerce « ses responsabilités en pleine indépendance » et que ses membres ne sollicitent ni n’acceptent « d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme ». Dès lors, comment rattacher la désignation de ses membres au pouvoir que l’exécutif exerce pour le bon fonctionnement de l’État ? Disons les choses autrement : le pouvoir de nomination, depuis l’âge classique, est l’une des plus importantes marques de souveraineté. L’exécutif en dispose, car, juridiquement, il dirige l’administration et, politiquement, il exerce une magistrature d’influence. Néanmoins, le commissaire européen incarne par hypothèse la délégation de souveraineté. Juridiquement et politiquement, il surplombe les États membres, contraint et concurrence leur activité législative et rivalise d’influence avec eux. Voilà d’ailleurs des décennies que la science politique décrit sa transformation progressive en véritable responsable politique au fur et à mesure que l’Union accumule les compétences. C’est pourquoi ranger à toute force le choix du commissaire dans les cases de l’article 13 de la Constitution pour conforter la prérogative présidentielle a quelque chose d’un peu paradoxal. Le refus opposé au Parlement de jeter ne serait ce qu’un regard sur ce choix est difficilement justifiable. La commission des affaires étrangères est donc reconnaissante au président Rapin de son initiative et de l’attention qu’il a prêtée à ses remarques au cours des travaux préparatoires. Ses amendements visent à clarifier la procédure et le format des auditions, mais aussi à expliciter le rôle des commissions compétentes pour les affaires étrangères dans l’audition du futur commissaire.

En effet, comme l’a très justement rappelé Mme Canayer dans son rapport pour la commission des lois, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions du 13 décembre 2012 et du 13 août 2015, « juge qu’en dehors de la procédure prévue par l’article 13 le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le pouvoir de nomination du Président de la République ou du Premier ministre soit subordonné même à la simple audition par le Parlement de la personne dont la nomination est envisagée Lorsque la France propose des candidats au sein de la Commission européenne, de la Cour de justice de Luxembourg ou de la Cour des comptes européenne, ces propositions sont assimilées, sans ambiguïté, à des nominations au sens et pour l’application de notre Constitution. Le fait que les désignations dont il s’agit ici relèvent de la conduite des relations internationales conforte encore le risque d’inconstitutionnalité du dispositif au regard des prérogatives de l’exécutif dans ce domaine. Les propositions d’amendements soumises depuis n’écartent aucunement cette difficulté. La jurisprudence est donc sans équivoque et devrait résonner en vous qui, en tant que parlementaires, êtes les défenseurs des institutions et du droit. À lui seul, le constat relatif au risque d’inconstitutionnalité du texte suffit à exclure le soutien du Gouvernement.

C’est en sens que le général de Gaulle affirmait lors du discours de Bayeux en 1946, dans le cadre de sa réflexion sur l’avenir de nos institutions, au lendemain de la libération de la France : « Il faut que l’autorité cesse d’être diluée et que le pouvoir exécutif puisse agir sans entrave dans son domaine propre. Tous les présidents, quelle que soit leur appartenance politique, ont depuis maintenu la spécificité de ce domaine réservé. Le renouvellement institutionnel de la Commission européenne, l’une des négociations les plus stratégiques l’échelon européen, relève indubitablement de la conduite de la politique étrangère et européenne de la Nation. En soumettant le pouvoir d’action du Président de la République à une audition parlementaire, cette proposition va à l’encontre de la philosophie qui a présidé jusqu’alors au fonctionnement

Par ailleurs, en projetant nos débats internes dans l’arène européenne et en exposant cette nomination au risque d’instrumentalisation politique, nous prendrions le risque d’affaiblir la voix de la France et de fragiliser le commissaire français. En effet, un candidat mis en cause ou désavoué par le Parlement national, quelles qu’en soient les raisons, risquerait de fragiliser notre posture dans ces négociations, où il importe d’afficher un front uni – ce qui, là encore,

agiter la France. Des exemples récents dans certains pays de l’Union européenne ont montré que l’instrumentalisation politique interne pouvait affaiblir le pays lors de la négociation du portefeuille. Le risque de politisation des nominations de juges à à la CJUE et de magistrats à la Cour des comptes européenne par le biais d’une audition parlementaire n’est pas non plus négligeable. Une politisation pourrait d’ailleurs constituer une entorse au principe d’indépendance et d’impartialité des candidats, comme certains d’entre vous l’ont bien noté. Le Gouvernement s’oppose donc également aux articles de la proposition de loi se rattachant à ces nominations.

autant, mesdames, messieurs les sénateurs, le risque d’inconstitutionnalité de l’intervention du Parlement dans les nominations, ainsi que son caractère inopportun, à notre sens, au regard des enjeux évoqués,

dans cette assemblée et à rendre, je l’espère, plus lisible pour nos concitoyens l’action européenne de la France. La réforme constitutionnelle de 2008 a également apporté son lot de progrès. Je pense à l’extension de la portée de l’article 88 4 de notre Constitution, qui conduit le Gouvernement à soumettre au Parlement, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets de réglementations Nous le savons, ce dispositif est perfectible, car il se heurte souvent au rythme législatif de Bruxelles. Toutefois, il vous revient d’en exploiter toutes les possibilités. Vous pouvez compter sur l’appui du Gouvernement en ce sens.

la disponibilité du Gouvernement pour échanger régulièrement sur les priorités européennes. Au delà du débat que nous aurons ce soir, je me tiens à votre disposition pour vous rendre des comptes

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, durant les premières décennies de leur construction, les institutions européennes ne passionnaient pas les foules. Aujourd’hui encore, il est souvent reproché à l’Union européenne d’être technocratique, voire déconnectée du réel, du quotidien et des préoccupations de nos concitoyens. Au fil des années, le rôle de l’Union européenne a été étendu. De crise en crise, les Européens ont été conduits à prendre conscience de l’impérieuse nécessité de s’unir plus étroitement. Les partis des extrêmes pouvaient encore, il y a quelques années, proposer de quitter l’Union européenne. Désormais, sans doute grâce au contre exemple du Brexit, plus personne n’est assez irréaliste pour prétendre qu’un pays européen, seul, pourrait faire face aux grandes puissances régionales du monde. L’invasion de l’Ukraine par Poutine, les manœuvres de Pékin ou encore l’inconstance de notre allié américain laissent au contraire penser que le renforcement du rôle de l’Union européenne devrait se poursuivre. À mesure que le pouvoir de ces instances s’accroît, notamment celui de la Commission européenne, les nominations deviennent de plus en plus stratégiques. Ce raisonnement a conduit le président Rapin à déposer la proposition de loi que nous examinons ce soir. Son objet est de renforcer la place du Parlement dans les nominations des candidats aux fonctions de commissaire européen, de membre de la Cour des comptes européenne ou encore de juge ou d’avocat général près les juridictions l’Union européenne. Le texte prévoit ainsi que les candidats pressentis seront auditionnés par les commissions du Parlement, auditions qui seraient suivies d’un vote consultatif. La perspective du renforcement des prérogatives du Parlement est toujours séduisante.

la rapporteure a toutefois indiqué en commission qu’il ne revenait pas à la commission des lois d’anticiper la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette position peut étonner lorsque l’on connaît la très grande sensibilité avec laquelle les commissions de notre assemblée appliquent les irrecevabilités au titre des articles 40 et 45 de la Constitution

L’inconstitutionnalité de ce texte devrait amplement suffire à provoquer son rejet. Nous devons cependant également examiner les conséquences que son adoption entraînerait. Le candidat resterait choisi par le pouvoir exécutif. Le Parlement serait consulté sans pouvoir s’opposer à sa nomination, mais il pourrait en revanche le désavouer.

À cet égard, même une absence d’unanimité pourrait suffire à éroder sa légitimité. Finalement, cette proposition de loi ne renforcerait aucunement la légitimité du candidat français, mais elle permettrait assurément au Parlement de l’affaiblir. Les divisions politiques intérieures sont une conséquence tout à fait normale de la démocratie ; en revanche, il nous semble que les afficher sur la scène internationale pourrait affaiblir la France. Quand bien même le Parlement verrait son pouvoir s’accroître, nous estimons qu’une telle réforme serait préjudiciable à notre pays. Pour que la France continue de peser au sein des institutions européennes, il nous paraît essentiel que les candidats français ne soient pas fragilisés.

permettre au Parlement national d’exercer un droit de regard sur la désignation des représentants français à des postes clés au sein des institutions européennes. texte s’inscrit pleinement dans le prolongement des réflexions menées au sein du groupe de travail transpartisan du Sénat sur les institutions, dont le rapport a été publié en mai 2024. Aujourd’hui, force est de constater que ces nominations, bien que stratégiques pour notre pays, sont décidées sans que le Parlement soit associé au processus. Cela a été particulièrement évident lors de la récente désignation du candidat français à la Commission européenne, intervenue dans des conditions qui ont soulevé de légitimes interrogations. Une telle situation ne peut plus perdurer si nous voulons restaurer la confiance de nos concitoyens dans nos institutions,

Cette proposition de loi vise ainsi à combler une lacune en instituant un mécanisme d’audition parlementaire préalable pour les candidats français à certaines fonctions européennes : commissaires européens, membres de la Cour des comptes européenne, juges et avocats à la Cour de justice de l’Union européenne et juges au tribunal de l’Union européenne. Ces auditions, qui seront ouvertes aux commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, garantiront un débat transparent et permettront d’évaluer les compétences et l’indépendance des candidats.

D’ailleurs, dix États membres de l’Union européenne associent déjà leurs parlements nationaux à la désignation de leurs commissaires européens, onze pays à celle des membres des juridictions européennes et neuf à celle des membres de la Cour des comptes européenne. Cette proposition de loi s’inscrit donc dans une véritable dynamique européenne de consolidation du rôle des parlements nationaux. La nomination des membres français des institutions européennes n’est pas une question purement purement formelle. Elle engage notre crédibilité collective et l’efficacité de ses représentants sur la scène européenne. En effet, comme le rappelle Jean François Rapin dans son exposé des motifs des motifs : « Cette nouvelle procédure permettrait d’évaluer les qualifications et l’expérience du candidat au regard des fonctions qu’il est appelé à exercer, mais aussi d’éclairer la représentation nationale sur les orientations que le candidat entend soutenir s’il est confirmé dans ses fonctions. » Ces nominations doivent être perçues non plus comme des décisions prises unilatéralement, mais bien comme un processus transparent et démocratique. La représentation nationale doit jouer pleinement son rôle en éclairant la pertinence des candidatures proposées par l’exécutif. Par ailleurs, cette initiative est cohérente avec l’esprit de la révision constitutionnelle de 2008, qui a renforcé le contrôle du Parlement sur certaines nominations nationales. Elle s’inscrit donc dans la même logique d’équilibre des pouvoirs, en permettant au Parlement d’exercer un contrôle démocratique sur des décisions qui engagent la place de la France en Europe. J’insiste, ce texte ne remet en cause ni les prérogatives de désignation de l’exécutif ni le domaine réservé du Président de la République. Monsieur le ministre, il s’agit non pas d’un droit de veto parlementaire, mais bien d’un outil au service de notre démocratie. Il permet d’associer le Parlement à des décisions cruciales tout en respectant les équilibres institutionnels. Il s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du rôle du Parlement dans les affaires européennes. Je sais que notre commission des affaires européennes y est particulièrement attachée. Ce pas supplémentaire permettrait d’associer étroitement les Français, leurs représentants, à des questions européennes d’une résonance majeure. C’est notre responsabilité, en particulier au regard des actualités géopolitiques, économiques, sociales et environnementales qui heurtent, parfois, les intérêts de la France et de l’Union européenne. Ainsi, en adoptant cette proposition de loi, le Sénat enverrait un signal fort en faveur d’un dialogue renouvelé entre les institutions européennes et les institutions nationales au sens large, d’une part, et leurs mandants – les Français –, d’autre part.

nous sommes saisis ce soir d’une initiative, louable, visant à renforcer l’influence de notre Parlement dans le jeu institutionnel européen. Vous conviendrez néanmoins que l’actualité, qui s’emballe, nous appelle à l’appréhender dans un contexte différent de celui qui a dû présider à sa gestation.

Dans ce contexte, nous sommes tous soucieux de préserver nos intérêts nationaux au sein de l’Union européenne et de garantir nos intérêts européens face à la véhémence des puissances expansionnistes, alors que l’Union est calomniée sur la place publique mondiale 64 % des Français s’inquiètent de la situation en Ukraine et des risques d’embrasement de l’Europe. Cette actualité brûlante nous appelle à faire bloc et à œuvrer avec pragmatisme pour préserver l’efficacité de notre propre influence dans le processus de décision bruxellois. Cette proposition de loi vise à rendre obligatoire une audition publique devant notre Parlement préalablement à certaines nominations au sein des institutions européennes, suivie d’un vote à caractère consultatif. Encore une fois, si cet objectif paraît louable, il convient de s’interroger sur les conséquences pratiques d’une telle mesure dans le contexte que nous connaissons. la nomination du commissaire européen, la consultation parlementaire préalable qui est souhaitée complexifiera sans équivoque notre processus de désignation. Or le droit de l’Union n’oblige aucunement les États membres à associer leur pouvoir législatif à cette sélection – cela a été rappelé.

Enfin, la comparaison des pratiques en vigueur dans certains autres États membres conduit à occulter la singularité du rôle joué au nom de la France par tous les chefs de l’État français, de gauche comme de droite, dans la construction de l’Europe depuis le début de ce grand dessein, au lendemain du dernier grand conflit mondial.

C’est le cas durant le processus de désignation par la voix du Conseil, où siège l’exécutif français ; lors de l’approbation du collège au Parlement européen, au sein duquel siègent les parlementaires français élus au suffrage universel direct ; enfin, lors de la nomination finale de la Commission par le Conseil. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, avec toute la considération et le respect que je porte, comme vous tous, à notre assemblée et au président Rapin, je m’interroge néanmoins sur l’opportunité de cette proposition de loi, dans le contexte mondial que nous connaissons. Faut il réellement engager une révision des règles de nomination en vigueur et remettre en cause par ce biais l’autorité du Président de la République française, au moment où la France doit tenir sa place et son rang au sein de l’Union européenne ? Faut il porter les joutes politiciennes et les divisions extrêmes, qui rongent notre Parlement depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, au sein des institutions européennes, à ce moment crucial de notre histoire ? Quelle sera notre capacité collective à désigner un candidat commun par la seule règle de la majorité dans les deux chambres, quand il nous a fallu trois gouvernements pour voter le budget de la Nation ? Mes chers collègues, la fonction présidentielle est essentielle en ces temps de tensions. N’alourdissons pas le navire quand il doit affronter la tempête

Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera contre cette proposition de loi. La parole

Historiquement, cette compétence se rattache à l’exercice du pouvoir exécutif. Les théoriciens de la souveraineté y ont même vu, à l’époque moderne, la prérogative royale la plus importante.

Dans la pratique, cette prérogative est le plus souvent restée la chasse gardée du Président de la République, et elle le restera si l’on en croit le discours que vient de tenir M. le ministre. La révision constitutionnelle de 2008 a pourtant amorcé une inflexion nécessaire en la matière. Depuis cette date, le Parlement auditionne les personnes nommées à une cinquantaine de fonctions jugées suffisamment importantes pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation. Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à élargir les prérogatives des chambres en soumettant à une audition les candidats pressentis aux postes de commissaire européen, de membre de la Cour des comptes européenne et aux fonctions de juge et d’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne concerne la désignation des candidats pressentis au poste de commissaire européen, nous partageons entièrement le raisonnement du président Rapin. Après l’épisode, pour le moins surprenant, de la démission de M. Thierry Breton en septembre dernier, il apparaît sain, pour notre compréhension de l’Union européenne et pour notre démocratie, aussi bien de clarifier les modes de nomination des commissaires français que d’auditionner les candidats pressentis à ces postes. Ces commissaires occupent en effet, comme vous le savez, une place essentielle au sein de l’exécutif européen. Que nous puissions auditionner le candidat français paraît donc, sur le principe, tout à fait raisonnable. De fait – cela a été rappelé –, de nombreux États en Europe ont déjà pris cette direction : dix parlements nationaux participent actuellement au processus de désignation de leur commissaire européen. En Autriche, le nom du candidat proposé fait même l’objet d’une véritable concertation entre les parlementaires et le gouvernement. Nous estimons que de telles auditions sont également souhaitables pour les candidats au poste de membre de la Cour des comptes européenne.

Sur ce point, je reste donc attachée au texte initial. Ce n’est pas nuire à l’indépendance des magistrats que d’avoir une conversation franche sur leur future fonction et la compréhension qu’ils en ont, en particulier lorsque ce vote n’est pas contraignant. D’ailleurs ces auditions sont pratiquées chez onze de nos voisins européens. En Allemagne, une commission spéciale est même désignée pour procéder à la nomination des juges allemands au sein du Tribunal et de la CJUE. Ces auditions, exactement comme celles qui sont prévues aux articles 1 et 2 de cette proposition de loi, permettraient surtout de mieux associer le Parlement aux désignations au sein de certaines institutions européennes particulièrement importantes. Enfin, je soutiendrai les amendements proposés par le président Rapin, qui visent à régler un certain nombre de difficultés soulevées par la rédaction initiale. Sans préjuger d’une éventuelle décision du Conseil constitutionnel, le groupe du RDSE votera ce texte, car il est essentiel pour l’avenir de l’Union européenne que les processus de désignation à ces postes clés soient mieux connus, plus transparents, et donc plus démocratiques. La

Le texte dont nous débattons aujourd’hui vise à renforcer le contrôle du Parlement dans le processus de désignation des candidats français à la Commission européenne, à la Cour des comptes européenne et aux juridictions européennes, en instaurant des auditions consultatives dans chaque assemblée parlementaire. Derrière ces dispositions se dessine clairement la volonté de parfaire la légitimité démocratique des institutions de l’Union européenne, une union dont les fondements demeurent les États souverains « unis dans la diversité ». C’est pourquoi il semble légitime que la représentation nationale, dont le Sénat, ait un droit de regard sur les propositions de nomination du Président de la République.

ne s’oppose en aucun cas aux actions du Parlement européen, elle est un complément ; elle enrichit donc la démarche de ce dernier. Oui, le Parlement national émet un avis sur les désignations proposées par le Président de la République, puis le Parlement européen est libre d’approuver ou non les candidatures ! Pourquoi ce droit accordé au Parlement européen serait il refusé aux parlements nationaux ?

Troisième objection : il existerait un risque d’inconstitutionnalité. Les rapporteurs vont nous soumettre des amendements visant à sécuriser le dispositif proposé, mais le risque existe bel et bien. Sur le plan purement juridique, seul le Conseil constitutionnel peut déclarer un texte législatif conforme à notre bloc de constitutionnalité ou le censurer. Sur le plan politique, je tiens à le préciser, bien qu’il soit vrai que les désignations pour les postes européens n’entrent pas dans le périmètre de l’article 13 de la Constitution, rien n’empêche, selon moi, la tenue d’un cycle d’auditions. Pour paraphraser les mots de la rapporteure Canayer, les désignations au poste de commissaire européen, notamment, relèvent d’une procédure ; il semble donc logique que le contrôle du Parlement national soit également. Pour conclure, il est essentiel de rappeler que nous étudions ce texte dans un contexte international inédit. À l’heure où nous assistons à un « basculement entre deux mondes », il nous faut plus d’Europe.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les élections européennes de juin 2024 ont marqué le début d’un nouveau cycle institutionnel pour l’Union européenne. Pourtant, la désignation du commissaire européen français s’est déroulée dans un climat particulièrement troublé. Alors que Thierry Breton était initialement pressenti pour siéger à la Commission européenne, il annonçait le 16 septembre dernier qu’il ne briguerait finalement pas ce poste.

La Commission européenne est composée de commissaires désignés par les États membres. Leur approbation relève du Parlement européen, non du bon vouloir de la présidente Cet épisode illustre une tendance lourde : l’effacement progressif de la souveraineté française au sein des institutions européennes, un processus enclenché dès la signature du traité de Maastricht. Il révèle surtout une réalité politique plus inquiétante : l’influence grandissante du capital allemand, dont l’industrie de défense est intrinsèquement liée à celle des États Unis, et qui impose de plus en plus ses choix stratégiques en Europe. Pourtant, face à cette mise en garde, le président Emmanuel Macron s’est empressé de s’aligner, en nommant Stéphane Séjourné sans la moindre résistance. la capacité de la France à défendre ses positions dans des secteurs aussi stratégiques que la défense, le nucléaire ou l’agriculture a été affaiblie. Ce texte vise justement, dans son article 1, à ce que le Parlement trouve toute sa place, au travers d’une consultation sur le choix du candidat proposé par le Président de la République pour le poste de commissaire européen.

Cependant, nous ne sommes pas favorables à l’idée d’accorder au Parlement un droit de regard sur la sélection des candidats aux postes de juge ou d’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne. en effet qu’une telle procédure porterait atteinte aux garanties d’indépendance dont le candidat doit bénéficier dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Selon nous, une telle audition parlementaire ferait peser le risque d’influences politiques, compromettant de fait l’impartialité requise pour ces fonctions. Malgré ce point, nous voterons ce texte, dont nous approuvons l’objectif de renforcement du rôle des parlements nationaux dans le processus de désignation des membres de certaines grandes institutions communautaires. nous tenons tout de même à affirmer que cette proposition de loi ne répond que très partiellement à l’enjeu de démocratisation de l’Union européenne. Pendant que nous débattons des modalités de nomination au sein des institutions européennes, un tournant majeur s’opère sur le continent l’Union européenne s’engage dans une reconfiguration profonde de sa politique de défense. Le président Macron appelle à augmenter les dépenses de défense pour les porter à 3 % ou 3,5 % du PIB. Qui assumera ce fardeau ?

redressement des finances publiques » et « nouvelles marges de manœuvre » face au contexte géopolitique. Autrement dit, le financement de cet effort reposera, une fois de plus, sur les travailleurs et les classes populaires. L’intérêt des peuples d’Europe ne réside certainement pas dans une surenchère militaire ou une intensification du conflit. Il s’agit non pas de nier la réalité des menaces, mais d’affirmer une autre voie. Tant que l’Union européenne continuera de fonctionner sur les mêmes bases, il ne pourra pas y avoir de véritable souveraineté démocratique. Tant que la Banque centrale européenne (BCE) restera hors de tout contrôle politique, tant que le marché intérieur sera conçu pour servir les intérêts des grands groupes pharmaceutiques, énergétiques et de l’armement, tant que la libéralisation sera un dogme, nous serons enfermés dans une logique qui nous échappe. Si la France veut véritablement peser au sein de l’Union européenne et retrouver la maîtrise de son destin, elle doit prendre l’initiative de rompre avec le pacte de stabilité et de croissance (PSC), mais pas pour alimenter un surarmement effréné ! Il faut rompre avec ce carcan budgétaire pour investir dans un autre modèle de développement, fondé sur le progrès humain et non sur une fuite en avant militariste. Investir dans l’avenir, c’est renforcer notre souveraineté industrielle, développer une industrie numérique publique et autonome,

les intérêts des marchés et des vendeurs de canons. Nous soutiendrons donc cette proposition de loi, mais nous continuerons à défendre une ambition bien plus grande : celle d’une rupture avec l’ordre maastrichtien et d’une refondation démocratique et sociale de l’Europe.

à protéger nos valeurs, l’État de droit et la confiance collective que nous avons dans nos institutions. L’incapacité de l’Europe à s’imposer aujourd’hui sur la scène internationale doit nous alerter non seulement sur notre sécurité militaire et sur notre poids diplomatique, mais aussi sur notre aptitude à prendre des décisions ensemble. Comment prétendre faire entendre une voix forte et sérieuse hors de nos murs, sans une Europe unifiée et cohérente à l’intérieur ? Il n’y aura pas d’Europe influente, respectée et capable sans des institutions plus intégrées, moins dépendantes de choix de connivence et du bon vouloir individuel de dirigeants nationaux. Renforcer l’Europe, cela doit se faire tant à l’échelle de l’Union qu’à celle des pays qui la composent. Aujourd’hui, en France,

Garantir que le Parlement puisse être consulté sur un choix aussi important fait, en son nom, par le Gouvernement n’est pas franchement extraordinaire, mais c’est un pas dans la bonne direction, un pas vers une responsabilisation renforcée de ceux qui nous représentent.

de la légitimité européenne dépasse très largement la seule question des nominations françaises dans le système existant. En ce qui concerne la Commission européenne, c’est le principe même de la nomination du collège des commissaires qu’il faudrait repenser.

qui nous a obligés à briser le tabou de la mutualisation des dettes publiques et qui a mis en évidence, une fois de plus, la toxicité de l’unanimité en matière budgétaire et fiscale. Nous le voyons avec la guerre en Ukraine, qui nous impose de développer une véritable défense européenne

de critères nationaux, c’est à dire d’un exécutif européen nommé, comme tout gouvernement, par la présidence de la Commission et élu par le Parlement européen.

C’est en suivant des utopies concrètes que nous avons maintenu la paix, si fragile, depuis soixante dix ans. Le trumpisme et le poutinisme ne sont pas dystopiques, ils existent réellement. La démocratie européenne,

vise à instituer la consultation préalable du Parlement sur la nomination de représentants de la France auprès de certaines institutions européennes. Sur le principe, nous ne pouvons qu’accueillir favorablement cette volonté de renforcer la place de nos assemblées dans le jeu institutionnel européen. ci est d’ailleurs conforme aux travaux transpartisans menés par le Sénat depuis plusieurs années afin de contribuer au nécessaire approfondissement démocratique du dialogue entre la représentation nationale et les institutions européennes.

nous l’avons indiqué lors de l’examen du texte en commission, nous émettons un certain nombre de réserves sur le cadre juridique et sur l’étendue des fonctions soumises à la consultation du Parlement.

Comme cela a été rappelé lors des précédentes interventions, si les procédures de nomination aux fonctions de commissaire européen, de membre de la Cour des comptes européenne et auprès du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne sont encadrées par les traités européens, le processus interne de sélection n’est cependant pas précisé. Les textes européens laissent en effet aux États membres la liberté de prévoir ou non des modalités de sélection des candidats envisagés pour occuper ces fonctions. À ce jour, le droit français n’a fixé aucune condition à ces désignations par les autorités, laissant place, il faut le dire, à une certaine opacité. la proposition de loi estiment nécessaire que la France s’aligne désormais sur les modalités mises en œuvre par plusieurs de nos partenaires européens, lesquelles prévoient une participation des parlements nationaux à la désignation des candidats aux

Cosac montrent qu’une minorité d’États ont instauré une participation de leurs parlements nationaux aux processus de nomination. Seule une dizaine des vingt sept États membres ont instauré un droit de regard de leurs parlements, selon des modalités extrêmement diverses.

sans pour autant explicitement avancer une proposition claire. Si la Cosac regrette que le renforcement du rôle des parlements nationaux ne figure pas parmi les priorités stratégiques de la nouvelle commission européenne,

lequel, nous l’avons dit, n’appelle pas d’objection particulière. Les modalités retenues par la minorité d’États membres ayant instauré ce droit de regard ne sont d’ailleurs pas uniformes. Cette proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, suscite pour cette Si le mode de désignation du commissaire européen mérite d’être encadré pour assurer une meilleure transparence, notamment au vu du caractère politique et stratégique de cette fonction, les modalités de la procédure envisagée à l’article 1 doivent être clarifiées. Les deux articles suivants relatifs aux désignations des candidats aux autres postes posent quant

à vous remercier

le commissaire européen sur proposition du Premier ministre interfère dans l’articulation entre les articles 13 et 21 de la Constitution, faisant courir un risque supplémentaire d’inconstitutionnalité. En pratique, bien sûr, le Président de la République et le Premier ministre s’entendent

le vote prévu par l’article 13 est un vote de validation. Il n’existe donc aucun obstacle à ce que la commission des affaires européennes vote à égalité avec une commission permanente. Il nous paraît

» les candidats aux priorités européennes du moment ou, pour le dire autrement, de tenter de soumettre le candidat à des injonctions politiques. À titre de comparaison, à l’échelon national, le Parlement n’est pas consulté sur la nomination des hauts magistrats tels que le vice président du Conseil d’État ou le premier président de la Cour de cassation. Par parallélisme, nous proposons de supprimer l’article